La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. En l’absence d’observations, je les considère comme adoptées.

ma collègue Amel Gacquerre a été enregistrée comme ne prenant pas part au vote alors qu’elle souhaitait voter pour. Acte vous est

celle ci préconisait de définir dans la loi des objectifs quantifiés et de réduire à 25 grammes par jour la consommation de sucre, pour chaque catégorie de produits. La surconsommation d’aliments industriels, notamment ultratransformés, favorise la survenance de maladies chroniques et, en particulier, une hausse régulière de la prévalence de l’obésité. D’après l’Inserm, les personnes obèses représentaient 8,5 % de la population en 1997 et 17 % en 2020. L’augmentation est encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes. Le nombre de cas d’obésité morbide,

la présence de sucres ajoutés en quantité importante par certains industriels qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle et de la nocivité de nombreux aliments transformés. Les maladies chroniques représentent pour nos sociétés un coût économique et financier considérable. Il est logique de reporter financièrement cette charge sur les industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop élevée. Il s’agit aussi de les inciter à proposer des produits plus vertueux et s’inscrivant dans le

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, M. Bonhomme l’a souligné, de 1997 à aujourd’hui, la proportion d’adultes en situation d’obésité ou de surpoids a doublé, passant de 8,5 % à 17 %, pour atteindre 9 millions de Français.

Cette information transparente et directe vise à mieux informer le consommateur dans ses achats et à inciter les industriels à améliorer la composition et la qualité nutritionnelle de leurs produits.

Je rappelle que le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents – cibles parfaites – fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel

comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité, notamment chez les plus jeunes. Certes, les programmes jeunesse font l’objet d’interdiction de publicité sur les chaînes publiques. Mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulation des professionnels demeurent trop timorées.

l’intermédiaire des influenceurs. Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants de moins de 16 ans, pour des denrées alimentaires nocives pour la santé.

haute teneur en alcool restent très disponibles à bas prix et bénéficient d’un fort appui publicitaire. C’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool à La Réunion doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance. Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques, d’une part, en vue de financer le fonds de lutte contre les addictions et, d’autre

en discussion commune,

Je vois bien que cela peut gêner certains. La commission est évidemment sensible à la situation évoquée par nos collègues ultramarins, mais elle ne peut être favorable à des amendements qui vont au rebours de tout objectif de santé publique.

qui a conduit à une augmentation moyenne de 70 centimes du paquet de cigarettes, à laquelle devrait s’ajouter une hausse de 40 centimes à 60 centimes au 1 janvier 2024. Pourtant, la récente hausse de la prévalence tabagique mesurée par Santé publique France devrait conduire les pouvoirs publics à repenser leur utilisation de la fiscalité comme principal outil de lutte contre le tabagisme. Le paquet de cigarettes le plus vendu a vu son prix passer de 7,5 euros en 2017 à 11,5 euros en 2023. Dans le même temps, le marché parallèle tout ce qui est consommé en France, mais qui n’a pas été acheté dans le réseau des buralistes – a explosé, et on estime désormais qu’il représente entre 20 % et 40 % de la consommation, alors que le réseau des buralistes est supposé assurer le monopole de la vente des produits du tabac. L’essor de ce marché parallèle a de graves conséquences en matière de santé publique, de lutte contre le tabagisme et de sécurité publique. La découverte de cinq usines de contrefaçon de cigarettes en quatorze mois sur le territoire français doit inviter les pouvoirs publics à réfléchir à une politique de santé qui ne reposerait pas essentiellement sur la pression fiscale, celle ci étant vigueur chez nos voisins européens. La surutilisation de l’outil fiscal devient contre productive et pousse les consommateurs à recourir à des stratégies de contournement, ce qui conduit au développement du marché parallèle. Ce phénomène est d’ailleurs accru dans le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat.

pour lutter contre la contrebande. J’étais à Charleville Mézières la semaine dernière. Je serai à la frontière espagnole vendredi. Notre priorité est de lutter de manière extrêmement résolue contre les trafics et la contrebande de tabac, qui ont lieu notamment dans les zones frontalières.

pour autant oublier ces millions de consommateurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas arrêter complètement de consommer du tabac ou de la nicotine. Cet amendement est donc

rapport, l’avis est toujours défavorable.

Ensuite, il est inexact de dire que le tabac à chauffer bénéficie d’un tarif préférentiel. La LFSS pour 2023, vous l’avez rappelé, a fixé une trajectoire fiscale de convergence avec les cigarettes, qui doit être achevée au 1 janvier 2026.

davantage maîtrisées : une politique de prévention est plus efficace et moins coûteuse pour notre système de santé que la prise en charge de l’ensemble des effets néfastes et secondaires découlant de la consommation de cannabis. Quel est l’avis de la commission ? Avis défavorable.

Ainsi, le budget publicitaire des plateformes a augmenté de 26 % entre 2019 et 2021. Ces campagnes publicitaires intensives incitent fortement des pratiques de jeu excessives. Aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60 % pour les paris sportifs.

En 2021, les opérateurs agréés sous droits exclusifs ont déclaré avoir investi 239 millions d’euros dans la publicité. Cependant, les jeux d’argent et de hasard provoquent des addictions puissantes, qui peuvent devenir incontrôlables et qui ont des conséquences sur la santé, comme sur la vie sociale, des personnes : surendettement et faillite, difficultés relationnelles et familiales, séparation, isolement professionnel, perte d’emploi, troubles psychologiques ou encore physiques, symptômes liés à la surconsommation associée d’alcool ou d’autres produits psychoactifs, dénutrition, suicide, etc. Ces campagnes de publicité visent par ailleurs un public très très jeune. La promesse est simple : l’enrichissement facile et rapide. Les opérateurs flirtent ainsi avec des lignes rouges, en menant des campagnes de communication qui reprennent les codes et le vocabulaire des quartiers populaires et des jeunes en particulier, en réalisant des publicités qui font miroiter une réussite sociale à travers le fait de gagner en pariant. Selon l’ANJ,

L’addiction aux jeux d’argent et de hasard est la seule addiction comportementale reconnue par l’OMS. Elle touche de plus en plus de jeunes, dont des mineurs, comme l’a montré une étude récente.

de parler en nous appuyant sur une réglementation plus stricte de la publicité sur les jeux d’argent et les paris sportifs en ligne.

Alimentée par le vieillissement de la population, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et une grappe d’innovations thérapeutiques, dont nous ne voyons pour le moment que les prémices, cette tendance devrait durer, voire s’accélérer. Alors que les difficultés d’approvisionnement s’accumulent chaque hiver, les enjeux sanitaires et de souveraineté que concentre le secteur sont par ailleurs évidents. Conçue comme une corde de rappel budgétaire par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 – cela ne date pas d’hier ! –, la clause de sauvegarde est devenue, depuis le milieu des années 2010, un véritable dispositif fiscal pesant sur les entreprises du médicament. Son poids a considérablement augmenté ces dernières années : alors que le rendement de la clause restait, depuis 2015, inférieur à 200 millions d’euros, il a atteint 1 milliard d’euros en 2022 et dépassera 1,5 milliard d’euros en 2023, comme en 2024. La clause de sauvegarde est ainsi devenue ces dernières années un outil de régulation des dépenses de médicament à part entière, comparable aux baisses de prix ou aux remises tarifaires négociées avec les industriels chaque année. que la commission l’a plusieurs fois souligné, la clause de sauvegarde ne fait pas un bon outil de régulation. Calculée l’année suivante dans le cas où les dépenses auraient dépassé le seuil prévu, elle est, d’abord, imprévisible pour les entreprises, qui se plaignent de l’incertitude dans laquelle elles sont placées.

Surtout, la clause étant répartie seulement en fonction du chiffre d’affaires des entreprises et de leur croissance, elle ne tient compte d’aucun impératif de santé publique ni d’aucun des enjeux industriels attachés à la production souveraine de médicaments. La commission a souhaité aborder cet article de manière pragmatique. Elle proposera de supprimer la réforme des modalités de liquidation de la clause de sauvegarde prévue par l’article 11. En effet, elle ne convainc pas les industriels et n’apporte aucune réponse aux écueils que j’ai décrits.

la priorité est au changement de nos rapports avec l’industrie pharmaceutique. La clause de sauvegarde a été conçue comme un mécanisme incitant à la négociation de prix dans le cadre d’une politique dite conventionnelle entre l’État et l’industrie pharmaceutique. Ce dispositif a été revendiqué comme un outil majeur de contrôle des prix. Le PLFSS 2024 vient non seulement relever le montant M, c’est à dire le plafond de dépenses à partir duquel la clause de sauvegarde sera déclenchée, mais aussi baisser la somme que les entreprises du médicament sont censées reverser à l’assurance maladie dans le cas où ce mécanisme serait déclenché. Ce relâchement du mécanisme de la clause de sauvegarde annonce une baisse de recettes pour l’assurance maladie sans contreparties transparentes, vérifiables et crédibles des entreprises de médicaments princeps sur les baisses des prix des innovations thérapeutiques. Si la clause de sauvegarde

efficacement au problème de régulation des prix des innovations thérapeutiques. La régulation doit passer par un plafonnement raisonnable des prix et des marges de profit de l’industrie. je propose que nous supprimions l’article 11 et que le Gouvernement commande un rapport indépendant sur la production d’un montant P fixant le seuil de profit des entreprises de médicament princeps. Quel

En faisant dépendre, à concurrence de 70 %, la contribution due par chaque entreprise de sa part dans le montant remboursé par l’assurance maladie, cette réforme concentre l’effort sur les industriels dont le portefeuille est composé de produits présentant un taux de prise en charge élevé. Tel est le cas des médicaments les plus indispensables à la prise en charge des patients : les médicaments dispensés en ville, qui présentent un service médical rendu important ; les médicaments innovants et onéreux dispensés à l’hôpital et pris en charge hors tarification à l’activité ; les médicaments intervenant dans le traitement d’une affection de longue durée. Cet effet est contraire aux préconisations de la récente commission d’enquête sénatoriale sur les pénuries de médicaments, qui invitait au contraire à mieux tenir compte de l’intérêt thérapeutique des médicaments et de leur criticité industrielle dans l’application de la clause de sauvegarde. La commission invite le Gouvernement à revoir cette réforme sans renoncer à l’objectif d’allégement des contraintes déclaratives pour les entreprises qu’elle entendait poursuivre.

La clause de sauvegarde est calculée au prorata de l’importance du niveau de dépassement du montant M. L’article 11, qui tend à réformer la clause de sauvegarde à partir de 2025, supprime la progressivité du calcul de la clause de sauvegarde et prévoit un taux unique de reversement à 90 %. Les travaux menés durant le premier semestre dans le cadre de la mission « Régulation des produits de santé », mandatée par la Première ministre, ont mis en avant la nécessité de remettre à plat la politique de régulation économique du médicament, notamment le fonctionnement de la clause de sauvegarde, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. En l’espèce, aucune analyse ni étude d’impact n’est fournie pour justifier l’augmentation du taux de reversement à 90 % à partir de 2025, alors même que le Gouvernement s’est engagé à stabiliser le niveau de régulation économique du médicament, qui a atteint des montants historiques entre 2021 et 2023. À cet égard, et à titre conservatoire, nous proposons de maintenir un taux unique de reversement à 70 %, dans l’attente de la présentation d’une étude d’impact permettant de réajuster ce taux de reversement à un niveau idoine.

de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche. Ce critère permettrait de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030, qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments, et dans l’esprit de la loi relative à l’industrie verte, qui vise une nouvelle étape de réindustrialisation du pays. Il permettrait également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et sur toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicaments.

11 prévoit d’aligner le fonctionnement du mécanisme de la clause de sauvegarde du médicament sur celui des dispositifs médicaux existant actuellement. Ainsi, le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde reposera non plus sur le chiffre d’affaires net déclaré par les entreprises, mais sur les montants nets remboursés par l’assurance maladie. La CGT estime que ce nouveau mode de calcul permettra aux grands groupes pharmaceutiques de réaliser des économies évaluées à 35 % de leurs bénéfices. Monsieur le ministre,

le plafonnement du montant dû par une entreprise au titre de la clause M à 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie, qui nous semble totalement injustifié. À titre d’exemple, au premier trimestre 2022, le laboratoire américain Pfizer a enregistré un chiffre d’affaires de 27 milliards de dollars, soit une hausse de 77 % en un an ; au premier trimestre 2020, Sanofi a publié un

nous paraît inapproprié, car il priverait la sécurité sociale de précieuses ressources. Nous l’avons vu depuis hier soir, la création de nouvelles recettes reste un tabou pour le Gouvernement, mais peut être n’est il pas nécessaire de supprimer ou de réduire celles qui existent…

vise à alléger la contribution au titre de la clause de sauvegarde des laboratoires exploitant des spécialités génériques, qui ont naturellement des marges

L’amendement n° 1328 rectifié vise à plafonner la contribution due par les entreprises au titre des médicaments génériques et médicaments de référence soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité qu’elles commercialisent à 2 % du chiffre d’affaires réalisé par ces médicaments. Il vise ainsi à mieux protéger ces médicaments du poids de la clause de sauvegarde. Le présent sous amendement a pour objet d’étendre le champ d’application des dispositions proposées en appliquant également le plafond de 2 % aux médicaments de référence dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à 5 euros, et ce même s’ils ne sont pas « génériqués ». Nous souhaitons ainsi mieux protéger du poids de la régulation l’ensemble des produits matures, peu onéreux et peu rentables, qui concentrent les difficultés d’approvisionnement observées ces dernières années.

du Comité économique des produits de santé (CEPS) le montant des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié pour les médicaments susceptibles d’être admis au remboursement, avant que le Conseil constitutionnel ne censure la disposition. Malgré un chiffre d’affaires en progression constante, l’industrie pharmaceutique critique depuis toujours cette clause de sauvegarde, en pointant le cas des génériques, initialement exclus du montant M. Les mécanismes de régulation des prix des médicaments viennent pallier l’absence de transparence dans la fixation des prix des médicaments,

tirée notamment par le vieillissement de la population, et à l’arrivée de nouveaux médicaments innovants, dont les prix sont souvent plus élevés, le présent amendement vise à garantir la neutralité financière, pour chaque entreprise, de la révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde.

L’objectif de cet amendement est de sécuriser et de préciser la procédure en introduisant cette disposition dans le texte relatif à la clause de sauvegarde. L’article R. 138 23 du code de la sécurité sociale étant d’ores et déjà appliqué, l’impact financier attendu de cette mesure est

visent à supprimer la réforme. Ainsi, nous entendons inviter le Gouvernement à la retravailler pour simplifier réellement les contraintes des entreprises et mieux tenir compte des enjeux de santé publique dans la clause de sauvegarde.

vise à étendre la mesure aux médicaments de référence dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à 5 euros et ainsi à limiter le poids de la régulation sur les médicaments matures les moins chers, qui concentrent les difficultés d’approvisionnement. Il s’agit d’une préconisation de la récente commission d’enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments.

des dépenses remboursées sur la liste en sus liées aux dispositifs médicaux, doit selon nous être revu dans son mécanisme. Aucun outil de pilotage ni aucune instruction de la part du ministère de la santé et de la prévention ou du ministère de l’économie n’existe ou n’est prévu à cette date pour anticiper un potentiel recouvrement de la clause. Si la hausse des dépenses en dispositifs médicaux à l’hôpital doit conduire à déclencher la clause de sauvegarde, il convient d’en étudier les facteurs, afin d’en tenir compte ultérieurement dans la méthodologie de calcul du montant Z d’apporter lisibilité et prévisibilité au secteur des dispositifs médicaux visé par l’obligation de contribution. Cette identification des facteurs de dépassement se justifie d’autant plus que la hausse du montant des dépenses remboursées n’est pas corrélée à

l’assurance maladie devra transmettre, dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de ce dépassement. Ce rapport devra permettre l’élaboration d’un outil de pilotage de la clause, mais également contribuer à la mise en place de mécanismes correctifs permettant de renforcer la prévisibilité et la stabilité de la régulation, ainsi que d’encourager l’émergence de l’innovation en France.

amendement vise à rendre applicables à la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux certaines des garanties envisagées dans le cadre de la réforme de la clause de sauvegarde des médicaments. Il tend notamment à préciser que l’assurance maladie et le CEPS doivent transmettre doivent transmettre à l’Acoss, avant le 15 juillet de l’année, les informations permettant la liquidation de la clause de sauvegarde. Ces informations seront transmises sans délai par l’Acoss aux entreprises concernées. Le retard accumulé dans la liquidation de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux pour 2022 est venu rappeler la nécessité de sécuriser la procédure de liquidation et d’améliorer la prévisibilité de la clause de sauvegarde pour les entreprises.

qui vise à encadrer la croissance, à l’hôpital, des dépenses remboursées sur la liste en sus liées aux dispositifs médicaux, doit être revu dans son mécanisme. En effet, le modèle de recouvrement de la clause, fondé sur un taux unique de contribution, apparaît comme un mécanisme dont la rigidité envoie un message fortement désincitatif pour la diffusion des produits de santé innovants en France. La situation est d’autant plus pénalisante que la hausse du montant des dépenses remboursées, dit « montant Z », n’est pas exclusivement corrélée à une surutilisation ou à un mésusage des dispositifs médicaux. Elle s’explique également par une évolution des besoins de santé dus à des changements organisationnels, comme le virage ambulatoire, sanitaires, comme la chronicité des maladies, ou encore technologiques, comme les prises en charge innovantes, que connaît le système de santé. Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir des aménagements circonstanciés de ce mécanisme pour, d’une part, assurer la prévisibilité et la stabilité de la régulation et, d’autre part, le rendre moins pénalisant pour l’émergence de l’innovation en France. Cet amendement vise donc à proposer une évolution du modèle de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux prenant en compte le risque accru de son déclenchement, afin d’introduire un barème de taux progressifs de contribution qui serait défini par voie réglementaire.

permet déjà de réduire le taux applicable à la part du montant remboursé excédant le montant Z, de 100 % à 90 %.

pour l’année 2023 pour tenir compte de l’incertitude pesant sur le secteur et de l’effet de rattrapage de son chiffre d’affaires après la crise sanitaire, le présent amendement vise à augmenter le montant Z pour 2024 en le portant à 2,45 milliards d’euros. Ce nouveau montant est obtenu en maintenant le taux d’évolution de 4,5 %, entre 2023 et 2024, retenu par le Gouvernement et en l’appliquant au montant Z pour 2023 rectifié permettra, le cas échéant, de maîtriser l’effet d’un déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux au titre de l’année 2024 et de mesurer les conséquences d’une telle taxation sur le secteur avant toute augmentation comparable à celle de la clause de sauvegarde des médicaments.

10 % de son chiffre d’affaires diminué des remises prises en compte dans le calcul de l’assiette de la clause de sauvegarde. Les entreprises du médicament, qui n’ont pas pris beaucoup de décisions d’amélioration de la prévention des risques de rupture de stock, doivent être mises à contribution pour participer à la solidarité de l’ensemble de notre système de santé. Cet amendement vise donc à supprimer la limitation du montant de la contribution due par chaque industriel du médicament à 10 % de son chiffre d’affaires. Quel

Un tel renforcement avait été soutenu par la commission en 2023. Il permet de maîtriser le poids de la clause de sauvegarde et de mieux tenir compte des efforts consentis par chaque entreprise. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. défavorable.

l’octroi de mer, la vie chère, les situations de quasi monopole, ou encore le nombre important de pharmacies rachetées par de grandes enseignes nationales, voire internationales. Tout cela fait que la majorité des officines achètent à flux tendu. Les stocks d’avance de ces médicaments sont donc localement insuffisants pour subvenir aux besoins des populations.

de la contribution sur vente de gros dans les collectivités ultramarines serait le bon moyen d’y répondre. Les effets d’une telle dérogation sur la constitution de stocks d’avance apparaissent en effet très incertains.

de produits de santé de la liste en sus, étape naturelle de régulation et de gestion de cette liste, suscitent toutefois un certain nombre de difficultés. En effet, établissements de santé, industriels, associations de patients et sociétés savantes ont récemment dénoncé, au travers d’un courrier adressé au ministre de la santé et de la prévention, le manque de concertation et d’anticipation des décisions de radiation survenues en fin d’année 2022, que l’impact de ces décisions sur les disparités d’accès aux soins, les pertes de chance pour les patients, les finances des hôpitaux publics et privés, ainsi que les surcoûts socio économiques liés au renoncement à ces thérapies. Ce constat, partagé par la Cour des comptes dans son rapport sur la tarification à l’activité de juin 2023, rend nécessaires des aménagements des procédures encadrant les radiations de la liste en sus, afin d’en renforcer la lisibilité et prévisibilité.

Ces rapports, remis aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la décision de radiation, doivent notamment permettre, lorsque cela est nécessaire, la mise en place de mécanismes correctifs

est également injuste du fait du seuil de 11 millions d’euros, qui induit une inégalité de traitement entre les acteurs économiques. Certains acteurs ont d’ailleurs scindé leurs activités, afin d’éviter cette taxe. La taxe est aussi sensible aux modes d’organisation de la distribution des produits par chaque société, disparité de traitement. C’est pourquoi il est proposé, par cet amendement, d’en simplifier le fonctionnement. Il est souhaitable de passer d’une taxe ne touchant qu’un petit nombre d’entreprises, avec un seuil aléatoire, à une contribution sur l’ensemble des entreprises

par la commercialisation de médicaments dérivés du plasma (MDP) issus d’un don non rémunéré et, d’autre part, le régime dérogatoire d’autorisation de mise sur le marché pour les produits dérivés du sang non conformes aux critères éthiques. Cette disposition va à l’encontre de la volonté de nos concitoyens, qui sont attachés aux valeurs humaines du don de l’Établissement français du sang (EFS), en matière de souveraineté sanitaire, en favorisant les laboratoires privés. Par cet amendement, nous voulons garantir l’indépendance nationale

comme tous les bénévoles, qui s’engagent fortement dans cet établissement. Destiné à produire des médicaments dérivés du sang, vitaux pour certains patients, le plasma doit faire face à une demande qui grimpe de 8 % par an dans le monde entier. La France, tout comme l’Europe, dépend à 65 % du plasma collecté aux États Unis, à partir de dons rémunérés. C’est pour réduire cette dépendance à 50 % que l’établissement a engagé en 2021 un plan Plasma pour 2026, avec un objectif de production à 1,4 million de litres Sur le plan éthique, l’enjeu est de pouvoir mieux répondre aux besoins des patients français, tout en préservant la sécurité des donneurs. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française pour le don de sang bénévole, qui nous alerte régulièrement. Quel

L’enjeu de sécurisation des approvisionnements en médicaments dérivés du plasma est récurrent. C’est pour limiter les vulnérabilités de la chaîne des approvisionnements que cet article vise à assouplir la législation française. Ensuite, l’article prévoit supprimer une exclusion de l’assiette de la contribution des entreprises pharmaceutiques sur le chiffre d’affaires correspondant aux médicaments dérivés du plasma. plasma. Il s’agit de remettre de l’équité entre tous les secteurs et les acteurs assujettis, sachant que le traitement particulier actuellement en vigueur s’accommode mal des exigences de l’Union européenne. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel est l’avis du Gouvernement ?

s’attache à défendre et promouvoir les valeurs du modèle français de collecte des produits du sang. Ce soutien se traduit d’ailleurs dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, par des dispositions qui seront discutées plus tard et qui visent à mettre en place un nouveau modèle de financement pour l’EFS. je le crois, attendu. Nous devons aussi aux patients l’accès aux médicaments dérivés du plasma. Or, aujourd’hui, les deux tiers de ces médicaments ne proviennent pas de la filière publique.

médicaux de 100 % à 90 % est nécessaire, notamment pour ne pas priver les entreprises de toute incitation à approvisionner la France lorsque le montant Z est dépassé. Cette disposition est soutenue par la commission, qui a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Poly, sur l’article. Selon l’article L. 131 7 du code de la sécurité sociale, « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale » donne lieu à « compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application ». Cette compensation intégrale s’interprète comme une compensation par crédits du budget de l’État, à l’euro, des pertes de recettes occasionnées pour la sécurité sociale. Toutefois, dans le cas des allégements généraux de cotisations sociales patronales, la compensation est réalisée par affectation de recettes fiscales. Par l’article 12, il s’agit d’approuver, pour 2024, la compensation de 7,1 milliards d’euros d’exonérations, réductions ou abattements de cotisations ou contributions de sécurité sociale. Ce montant est en augmentation par rapport aux années précédentes : +500 millions d’euros par rapport à 2022, et +1,7 milliard d’euros par rapport à 2021. Il ne couvre pas l’intégralité des exonérations de cotisations sociales. En effet, en 2024, l’État ne compensera

et continuerons de dénoncer ces mécanismes d’exonérations de cotisations, dans lesquels la sécurité sociale se retrouve doublement perdante, avec des cotisations patronales moindres, qui ne sont pas compensées par le budget de l’État. L’amendement

donc insuffisante, à la sécurité sociale du coût des exonérations de cotisations sociales. Les exonérations de cotisations sociales ne cessent d’augmenter, au point que, selon le rapport Ferracci et Guedj, les cotisations représentent aujourd’hui seulement 49 % des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale,

d’euros à la sécurité sociale pour l’exercice 2024. Les mesures non compensées que vous avez évoquées demeurent une exception. Elles se justifient à chaque fois par un partage de l’effort entre l’État et la sécurité sociale

l’inflation et les dépenses d’investissement. La Fédération hospitalière de France (FHF) estime qu’un abondement de 2 milliards d’euros est nécessaire pour 2024. On a longtemps considéré qu’il faudrait – toutes choses égales par ailleurs, c’est à dire sans les réformes profondes

pour tenir compte du vieillissement de la population, des innovations et de la croissance des pathologies chroniques. Ce PLFSS s’inscrit donc dans une trajectoire d’austérité,

La société de la protection de la pleine santé que les écologistes appellent de leurs vœux demande deux grands mouvements : sortir de la logique de l’enveloppe budgétaire fermée, pour passer à une logique d’investissements pluriannuels, à partir d’une analyse des besoins, notamment territoriaux ; en finir avec le cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique. Les décisions budgétaires reproduisent en fait les inégalités sociales de santé. Les personnes les plus précaires ont trois fois plus de risques de renoncer aux soins que les autres, les 10 % les plus précaires consacrent 7,5 % de leurs revenus à leur santé, contre 2,4

des dépenses de santé, estimée à 4 % par la commission des comptes de la sécurité sociale. Par rapport à l’évolution « naturelle » des dépenses, le Gouvernement compresse les dépenses de santé à hauteur de 1,5 milliard d’euros environ. Si on tient compte de l’inflation, la hausse de l’Ondam sera marginale. Le Gouvernement prévoit de réaliser par ailleurs 3,5 milliards d’euros d’économies, notamment sur les dépenses de soins de ville, la régulation des dépenses de médicaments et la hausse du ticket modérateur en dentaire, à hauteur de 500 millions d’euros à la charge des complémentaires santé. Le Gouvernement prévoit de réaliser 500 millions d’euros d’économies sur l’hôpital au nom de l’efficience. La Fédération hospitalière de France a d’ailleurs sommé le Gouvernement de « dire franchement ce qu’il souhaite » pour les hôpitaux publics, en pointant le décalage entre les annonces de refinancement de l’hôpital public et le budget de l’assurance maladie pour 2024. Les dépenses hors personnels augmentent de l’ordre de 15 % et les hôpitaux subissent un effet report de la hausse des prix de l’énergie. La dégradation de la situation financière des hôpitaux est d’autant plus préoccupante qu’elle pèse sur leur capacité à investir. Selon la Fédération hospitalière de France, il manque 1,9 milliard d’euros pour l’hôpital au titre de 2023 et 2 milliards d’euros au de 2024. La situation n’est pas plus réjouissante pour la médecine de ville, puisque le sous objectif de l’Ondam relatif aux soins de ville progresse seulement de alors que le territoire national est un gigantesque désert médical. Pour l’ensemble de ces raisons, nous refusons cet Ondam, largement insuffisant pour répondre aux besoins, et nous demandons la suppression de cet article. La

sous évalué, ce qui contraint dangereusement les réponses aux besoins sanitaires et sociaux de notre pays. La Fédération hospitalière de France estime qu’il faudrait que l’Ondam évolue globalement de 5,1 milliards d’euros. Nous croyons que ces tableaux ne reflètent pas la réalité des comptes sociaux et que tous les périmètres de la comptabilité nationale ne sont pas pris en considération. En effet, alors que la sécurité sociale était quasiment à l’équilibre en 2017, elle aura un déficit de 12 milliards d’euros en 2024 et de 20 milliards en 2027. en 2027. Cet appauvrissement de notre bien commun qu’est la sécurité sociale va à l’encontre des besoins sanitaires et sociaux, qui ne font que croître. Le Gouvernement, en sous évaluant l’Ondam, organise l’incapacité chronique de la sécurité sociale à répondre aux grands défis de la santé

démographique croît, et aucune réponse n’est apportée. L’accès aux soins pour tous est compromis pour nombre de nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article, traduction chiffrée de choix politiques auxquels nous sommes farouchement opposés.

2022. Je comprends que vous soyez opposés aux prévisions que traduisent ces tableaux d’équilibre pour 2024, et j’ai bien entendu les raisons pour lesquelles vous voulez supprimer cet article obligatoire.

pour couvrir les charges d’inflation, à hauteur de 800 millions d’euros. Les établissements ont bénéficié d’un bouclier énergétique évalué à 300 millions d’euros. Pour autant,

en hausse en 2024 de 1,4 milliard d’euros. Cet effort s’adresse à la fois aux familles des classes moyennes et aux plus vulnérables. La branche famille couvre en effet 13,7 millions de familles, et le plafond de ressources pour les allocations familiales à taux plein est de 71 000 euros pour un couple avec deux enfants.

La réalité a été rappelée par nos collègues, en particulier Annie Le Houerou. Nous ne pouvons pas approuver un tableau d’équilibre par branches pour 2024

ou,, précipiter sa perte ? Les cinq fédérations hospitalières expliquent qu’il manque 1,5 milliard d’euros simplement pour faire face au coût de l’inflation. Vous évoquez un financement spécifique de 800 millions d’euros ; c’est à peine la moitié. Le déficit des hôpitaux publics a doublé entre 2019 et 2022. Sur l’autonomie, 80 % des Ehpad

Durant la pandémie de covid 19, le gouvernement d’Emmanuel Macron a fait le choix de faire peser les 150 milliards d’euros de dette covid sur la Caisse En 2020, la majorité du Sénat avait critiqué le choix de transférer la prise en charge de la dette covid des caisses de l’État en prolongeant l’existence de la Cades de 2033 jusqu’en 2044. Avec la Cades, le Gouvernement impose à la sécurité sociale de passer par les marchés financiers pour refinancer sa dette. L’amortissement de la dette sociale pèse lourdement sur les comptes de la sécurité sociale. Se passer de 16 milliards d’euros signifie se tirer une balle dans le pied alors que nous avons besoin d’investir aujourd’hui dans la formation des professionnels de santé, paramédicaux ou sociaux, et de revaloriser les conditions de travail des aides à domicile. C’est aujourd’hui que nous avons besoin d’investir dans notre système hospitalier. C’est aujourd’hui que nous devons maintenir ouvertes nos maternités. Lorsque les services des urgences seront fermés les week ends et les soirs, les économies réalisées aujourd’hui entraîneront demain des coûts largement supérieurs.

Un transfert de déficit à hauteur de 136 milliards d’euros a été voté en 2020 ; il reprenait les déficits antérieurs, ainsi que les déficits des exercices 2020 à 2023 résultant de la crise sanitaire. Des recettes à hauteur de 16 milliards d’euros en 2024 ont été affectées à la Cades, afin d’assurer le remboursement de ces transferts, remboursement qui est prévu au plus tard pour 2033. 2033. Supprimer ces recettes serait contraire à la loi organique de 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et priverait concrètement la sécurité sociale d’un gage de soutenabilité et de pérennité ; je ne pense pas que cela soit votre objectif. Par ailleurs, affecter ces recettes à des dépenses nouvelles

Actuellement, la dette de la sécurité sociale est placée sur les marchés financiers. La solidité de notre modèle de protection sociale de presque quatre vingts ans est reconnue, y compris par par les établissements bancaires, puisque l’agence de notation Standard & Poor’s a donné la note la plus élevée en 2022 aux titres financiers de l’Acoss. Les établissements financiers se disputent les créances de la sécurité sociale, que l’on nous présente comme un spectre dangereux. La dette de la sécurité sociale est détenue par des établissements financiers dont nous ne connaissons pas l’identité, ce qui pose une difficulté en matière de souveraineté nationale. Surtout, et c’est l’objet de cet amendement, la dette de la sécurité sociale est détenue par des établissements enregistrés dans des paradis fiscaux. Cette réalité est d’autant plus choquante que notre modèle de protection sociale

En effet, alors qu’après la crise des dettes souveraines le déficit des Robss avait été réduit de manière continue de 2011 à 2019, l’Ondam ayant alors toujours été respecté, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale ne prévoit même pas de stabiliser le déficit, qui passerait de 8,8 milliards d’euros

et suppose une croissance de l’Ondam d’environ 3 % par an, alors que l’Ondam n’a plus été respecté depuis 2020, avec, en 2023, une croissance de l’Ondam de 4,8 % hors dépenses de crise et un dépassement estimé à 3,5 milliards d’euros par rapport à la

Oui, nous avons besoin d’une vision à long terme du financement de la sécurité sociale et d’une programmation pluriannuelle en matière de santé et de social. C’était d’ailleurs l’objet de l’un de mes amendements – jugé irrecevable –, ce qui devrait être acté dans une loi organique. En tout cas, c’est une proposition que je vous soumets. Mais non, cette prévision n’est pas soutenable ou réaliste. Le Gouvernement considère ainsi une prévision de croissance de 1,4 %, supérieure à celle du consensus des économistes établie à 0,8 %. Il prévoit un déficit croissant de la sécurité sociale sur des hypothèses d’inflation optimistes ; c’est dire Je ne m’épanche pas davantage sur les éléments financiers contenus dans l’avis du Haut Conseil des finances publiques. De plus, cette prévision n’entame aucun virage écologique ou d’investissement massif pour notre santé. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 16.

pluriannuelle du financement de la sécurité sociale pour les années 2023 à 2027. Le Gouvernement s’est engagé envers Bruxelles à limiter la hausse des dépenses publiques à 0,6 % par pour contenir les déficits en dessous des 3 %. Les dépenses de l’assurance maladie qui progressent seulement de 3,2 % cette année sont plafonnées à 3 % en 2025 et à 2,9 en 2026. Cette trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base est en total décalage avec la crise des hôpitaux, les difficultés des acteurs de santé et les besoins pour l’accompagnement de nos aînés, ainsi que pour améliorer la prise en charge des familles et des personnes en situation de handicap. De plus, la branche vieillesse voit son excédent se creuser à 14 milliards d’euros en 2027, ce qui suffit à montrer toute l’inefficacité de la réforme des retraites imposée au pays. Pour mémoire, le Conseil d’orientation des retraites estimait avant votre réforme que le déficit en 2027 se situerait entre 7,5 milliards d’euros et 10 milliards d’euros. Vous avez donc ajouté deux années de travail et une année de cotisation à l’ensemble des salariés au nom de l’équilibre du système de retraite pour finalement doubler le déficit prévu en 2027. Exactement ! Vos choix politiques sont contre productifs. Nous ne sommes pas les seuls à le penser dans ce pays. Je songe notamment aux organisations syndicales.

l’ampleur des cotisations à prélever. Ce débat est interdit au motif que la seule piste à

17,1 milliards en 2026., si cette dette n’était pas intégrée, les administrations de sécurité sociale dégageraient un fort excédent de 0,5 point de PIB en 2022 et 0,8 point

d’augmenter le taux de la contribution sociale généralisée sur les produits de patrimoine et les produits de placement ; de renforcer la taxation des retraites chapeaux des dirigeants des grandes entreprises ; d’augmenter le taux de cotisation des stock options et des actions gratuites ; d’augmenter le taux de forfait social sur les plans d’épargne de retraite, l’intéressement et la participation ; d’augmenter la contribution des employeurs ; d’instituer une contribution de solidarité des actionnaires d’instituer une contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des super profits ; d’instituer une contribution des revenus financiers ; d’instituer une contribution sur les revenus des Ehpad privés à but lucratif ; de supprimer

pluriannuelle des dépenses de l’assurance maladie conformément aux recommandations de la mission régulation des produits de santé. Il vise à articuler l’objectif salutaire d’une planification des dépenses sur une base triennale, avec la mise en œuvre d’une régulation basée, elle aussi, sur un cadre triennal. Cela permet donc d’intégrer pleinement les recommandations de la mission des produits de santé, en assurant leur traduction dans l’ordre juridique dès l’année 2024.

alinéa 2, du règlement, si le Sénat n’adopte pas les dispositions de cette partie, la troisième partie du projet de loi sera considérée comme rejetée. Y a t il des demandes d’explication de vote ?…

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

sociale visent à renforcer le volet prévention en y allouant 150 millions d’euros supplémentaires. Cela permettra la généralisation de la vaccination contre les infections à papillomavirus, la prise en charge intégrale des protections périodiques réutilisables pour les moins de 26 ans, la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 26 ans et l’évolution des modalités d’organisation des rendez vous de prévention aux âges clés. Il est nécessaire d’engager un véritable changement culturel sur le sujet, car la prévention permet une meilleure prise en charge des pathologies et un coût plus faible pour l’assurance maladie. Certains critiqueront le coût élevé de la prévention ; c’est une vision à court terme. La prévention est un investissement sur le long terme, car elle permet d’anticiper des maux nouveaux, dont le soin demanderait un budget plus important que celui de la prévention. Par un suivi régulier tout au long de la vie dès le plus jeune âge, chaque Français peut ainsi préserver sa santé et la soutenabilité de notre système de soins. sur l’article. Cet article 17 concerne le financement de la campagne de vaccination contre le papillomavirus, qui entraîne 6 400 cas de cancer par an, dont 3 000 cancers du col de l’utérus. Cette vaccination prévient 90 % des infections, voire 100 % si elle est pratiquée en début d’activités sexuelles. En France, la vaccination est recommandée depuis 2007 pour les jeunes filles et depuis 2019 pour les garçons de 11 ans à 14 ans et de 15 ans à 19 ans. La couverture vaccinale s’améliore depuis quelques années, mais demeure très insuffisante, avec 41 % chez les filles et 8 % pour les garçons. L’objectif

je salue les dispositions de l’article 17 relatives à la mise en œuvre de la vaccination HPV dans les collèges. Celles ci devraient permettre de rattraper notre retard et de protéger mieux l’avenir des filles et des garçons.

des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé. La fixation des tarifs des vacations pour la vaccination contre les HPV ne doit pas se faire sans les professionnels de santé. La dérogation au champ conventionnel devient trop habituelle, et c’est regrettable. Rien que dans ce PLFSS, plusieurs articles prévoient d’y déroger. Je pense notamment à l’article 20 – nous y reviendrons. Néanmoins, la dérogation me semble ici pouvoir être entendue, compte tenu du déploiement déjà engagé de la campagne de vaccination et de la diversité des professionnels de santé qui seront mobilisés, non seulement les professionnels libéraux, mais aussi les professionnels salariés intervenant en dehors de leur cadre habituel, ainsi que les étudiants. Dans ce contexte, l’ouverture de discussions conventionnelles apparaît complexe. la consultation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé est indispensable sur ce sujet, qui aurait dû faire l’objet d’une concertation préalable. C’est une garantie minimale de dialogue, qui ne doit pas être qu’un accessoire à la politique du Gouvernement. Quel est l’avis du Gouvernement

Je comprends parfaitement le raisonnement de Mme la rapporteure. Mais, pour trois séries de raisons, je considère que ce qu’elle propose

Et, comme on l’a vu, par exemple, pour les médecins en début d’année, cette négociation peut échouer. Si l’on renvoie à la négociation conventionnelle la fixation des tarifs d’une campagne de vaccination,

avec tous les professionnels de santé qui vont être habilités à vacciner, ce qui pose une difficulté encore plus importante, puisqu’il n’existe pas, dans le code de la sécurité sociale, de dispositions qui permettent

et que cette démarche d’« aller vers » soit bénéfique, il est nécessaire de prévoir des actions d’information efficaces dans les collèges et les établissements sociaux et médico sociaux concernés, pour permettre aux enfants et à leurs familles de prendre des décisions éclairées quant à cette vaccination. Tel

La vaccination contre le papillomavirus humain permet de prévenir les infections par les papillomavirus responsables de 70 % à 90 % des cancers du col de l’utérus. Le vaccin contre les infections à papillomavirus humain est la cible de nombreuses critiques, liées à une campagne de désinformation massive, comme l’a rappelé M. Chasseing. Cela s’accompagne d’une présence de mouvements antivax dans les médias, qui suscitent une méfiance généralisée envers la vaccination dans la population générale. Nous devons regagner

pour le permettre. En ce sens, la prévention du cancer du col de l’utérus ne doit pas être laissée aux joutes politiques et ne doit pas représenter un combat idéologique, au profit d’une vision conservatrice de la sexualité. La prévention du cancer doit primer sur toute considération sociopolitique ou religieuse, quelle qu’elle soit.

observés. Si des symptômes graves, comme le syndrome de Guillain Barré, ont pu être signalés, ils restent extrêmement rares. Des temps de sensibilisation et d’information doivent être organisés en amont des campagnes de vaccination auprès des élèves et de leurs familles, afin d’inciter le plus d’enfants, d’adolescents et d’adolescentes à se faire vacciner. La sensibilisation a été jugée irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. J’invite le Gouvernement à lever le gage. L’amendement

dans la grande partie des cas, ces infections disparaissent de manière naturelle, elles peuvent persister et évoluer vers des cancers. En France, 6 400 nouveaux cas de cancer sont ainsi causés, chaque année, par les infections HPV.

elle est retenue en Savoie en raison de problèmes liés aux inondations. Cet amendement vise à ce que le calendrier des vaccinations soit mis à jour régulièrement, dès la publication de nouveaux avis de la Haute Autorité de santé (HAS), afin d’assurer une meilleure prise en charge des personnes à risques dans les délais adéquats.

Gouvernement ? Madame la sénatrice, la HAS publie, chaque année, au moment de la semaine de la vaccination – au cours du premier trimestre –, son calendrier de vaccination.

: La parole est à Mme Anne Souyris. L’article 17 est prometteur sur la réalisation d’un rapport qui analysera l’opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humain dans des lieux qui ne relèvent pas de l’éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture. Cependant, les établissements scolaires privés sous contrat restent les parents pauvres de la politique de prévention scolaire. Certains établissements privés sous contrat, notamment ceux qui sont rattachés à une appartenance religieuse, peuvent être quant à l’organisation d’une campagne de vaccination HPV, en ce qu’elle se rattache à l’éducation sexuelle des plus jeunes. L’information des enfants, des adolescentes et des adolescents et de leurs familles doit primer sur des considérations politiques et religieuses. Nous avons besoin d’un rapport qui déterminera les modalités permettant de rendre

Cet amendement vise à compléter les sujets sur lesquels porte le rapport d’évaluation prévu par le présent article, en y inscrivant une évaluation de la campagne de vaccination dans les établissements privés et une réflexion sur la possibilité de rendre obligatoires les campagnes de vaccination dans ces établissements. En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité de la campagne de vaccination, celle ci entre déjà dans le champ de l’article. Pour ce qui relève d’une réflexion sur une obligation de déploiement de la vaccination dans ces établissements, il faut d’abord indiquer que les établissements privés peuvent tout à fait participer à la campagne de vaccination. En revanche, imposer celle ci pourrait susciter plus d’opposition que d’adhésion. Cette mesure pourrait malencontreusement être assimilée à l’obligation vaccinale, ce qui aurait un effet contre productif. en matière de vaccination, il faut agir par la pédagogie pour emporter la conviction de tous. Il revient néanmoins au Gouvernement d’œuvrer pour faire en sorte qu’un maximum d’établissements privés sous contrat acceptent de participer à cette première campagne et à celles qui suivront. Enfin, rien n’interdit aux parents d’adolescents scolarisés dans un établissement privé de recourir à cette vaccination en dehors du cadre scolaire. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel est

parole est à Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à clarifier les règles de vaccination contre les méningocoques. Compte tenu d’une recrudescence des infections invasives à méningocoques, la Haute Autorité de santé a été saisie en avril 2023 pour avis sur l’actualisation de la stratégie de vaccination. En effet, à ce jour, le code de la santé publique prévoit uniquement la vaccination obligatoire contre le méningocoque de sérogroupe C. L’amendement tend à permettre d’étendre, par voie de décret en Conseil d’État, l’obligation de vaccination contre les autres sérogroupes qui seront concernés, le cas échéant, par les recommandations de la HAS. Il a également pour objet d’actualiser le dispositif de suivi de la réforme de 2018 sur l’extension des obligations vaccinales des nourrissons. Quel

? Je considère que l’amendement, tel qu’il est proposé, répond à une vraie question de santé publique. En effet, on constate une recrudescence des infections invasives à méningocoques sur les sérogroupes A, C, W et Y,

été déposé sur l’initiative de Marie Do Aeschlimann. Bien que moins connus que leurs homologues masculins, les préservatifs féminins jouent un rôle crucial, tant dans la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) que dans l’autonomisation sexuelle des femmes. Cette dernière est d’autant plus pertinente face à l’augmentation des cas de, pratique consistant à retirer un préservatif masculin sans consentement pendant un rapport sexuel. Actuellement, l’utilisation limitée des préservatifs féminins peut être attribuée à leur coût élevé – environ 9 euros pour trois unités. Pour pallier ce problème, cet amendement vise à étendre le remboursement non seulement aux préservatifs masculins, mais aussi aux préservatifs féminins. L’objectif est d’inscrire ces derniers sur la liste des produits remboursables selon l’article L. 165 1 du code de la sécurité sociale. Cette proposition s’aligne, en outre, avec l’annonce faite par Mme la Première ministre le 8 mars dernier, visant à rendre les préservatifs féminins gratuitement accessibles sans ordonnance jusqu’à l’âge de 25 ans. L’adoption de cet amendement constituerait une étape significative vers l’égalité des sexes en matière de protection sanitaire et de contrôle sur la santé sexuelle.

Je précise cependant que « interne » et « externe » n’est pas une nouvelle façon de dire « féminin » et « masculin », puisqu’il y a des préservatifs internes à destination des hommes.

: La parole est à Mme Anne Souyris. Les associations de lutte contre la précarité menstruelle et de promotion de la santé menstruelle connaissent mieux que nous les enjeux sociaux et environnementaux de la santé menstruelle. Ce sont elles qui ont contribué à révéler la présence de composés toxiques dans les serviettes hygiéniques. Ce sont elles qui ont appelé à davantage de transparence dans la composition de ces produits. Ce sont elles, enfin, qui ont dénoncé la TVA honteuse à 20 % sur les protections menstruelles, abaissée depuis au taux de 5,5 %. Intégrer les associations expertes en santé menstruelle au processus de définition des critères de référencement des protections menstruelles réutilisables prises en charge par la sécurité sociale est indispensable pour

En conséquence, les prérequis à la fois techniques et de transparence sont garantis dans cette procédure. Les associations de promotion de la santé menstruelle pourront faire valoir des demandes, ce qui est leur rôle, mais il ne semble pas opportun d’inscrire une obligation de concertation avec lesdites associations dans le cadre de cette procédure. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable. Quel est l’avis du Gouvernement ?

la santé menstruelle au travail demeure largement ignorée. Alors que la moitié des femmes souffrent de dysménorrhée et qu’une sur dix est touchée par l’endométriose, cette question demeure relativement invisibilisée en France. Ce sujet est encore l’objet d’un tabou dans notre pays, alors que le Japon, l’Indonésie, la Corée du Sud ou Taïwan ont déjà adopté la création d’un d’un congé menstruel depuis plusieurs décennies, répondant ainsi à cet impératif de santé publique et de bien être au travail. Depuis février 2023, l’Espagne est le premier pays européen à leur avoir emboîté le pas. En France, des entreprises et des collectivités montrent la voie, à l’instar de Saint Ouen sur Seine, en Seine Saint Denis,

vue d’étudier l’opportunité de supprimer l’âge limite de la prise en charge des protections périodiques menstruelles pour les femmes de plus de 26 ans. En effet, la précarité menstruelle ne s’arrête pas à 26 ans.

La prévention en santé mentale est une nécessité pour remédier à la crise de l’offre de soins en santé mentale et en psychiatrie. Une attention toute particulière doit être portée à la pédopsychiatrie et à la détection précoce des pathologies lors des consultations de prévention. Quel